J'ai mal à ma France » a twitté Kylian Mbappé, disant avec ses mots ce que ressentent des millions de jeunes et de parents, choqués par la vidéo du drame. On y voit un policier braquer son arme à bout portant par la portière du véhicule et tirer mortellement sur le conducteur, un jeune de 17 ans. Je pense que cette émotion est également présente dans les commissariats de France, où les fonctionnaires sont nombreux, ce matin, à avoir mal à leur métier.

Je dis ma solidarité à la famille du jeune Nahel. Je dis également mon soutien entier au maire de Nanterre, Patrick Jarry, et aux élus de cette grande ville populaire, qui veulent la vérité. La vidéo du contrôle et du tir est glaçante. Le policier a été placé en garde de vue et mis en examen pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. C'est dire la gravité des faits soumis désormais à enquête.

Au-delà de cette enquête, qui doit suivre son cours rapidement, est-il envisagé, madame la Première ministre, afin de réagir à la mesure des faits incriminés, de prononcer une suspension à titre conservatoire de l'agent concerné ?

Madame la Première ministre, un pays dans lequel la police et la jeunesse ne peuvent se croiser sans inquiétude et angoisse est un pays malade de sa démocratie. Il relève de votre responsabilité de changer au plus vite ce climat.

hier, à Nanterre, lors d'un contrôle routier, un jeune homme de 17 ans a été tué. C'est un terrible drame. Je veux commencer par dire ma profonde émotion et par adresser mes condoléances à sa famille, à ses proches et à ceux de son quartier. Le Président de la République a eu l'occasion de le rappeler ce matin : c'est la Nation tout entière qui est touchée par ce drame. Je me suis entretenue avec le maire de Nanterre, Patrick Jarry. Je lui ai dit mon soutien et celui de mon gouvernement. ai fait part de notre détermination à ce que toute la vérité soit faite. Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil et une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes, au quotidien, sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice devra établir les faits. Elle a été saisie et a commencé son travail : un policier est en garde à vue. Je souhaite comme chacun que la vérité soit faite le plus rapidement possible et que des réponses soient apportées. La justice passera, personne ne doit en douter. Seule la justice permettra de faire toute la lumière sur ce drame. Seule la justice apportera des réponses face à la douleur d'une famille et à la peine d'une nation. Seule la justice garantira notre unité. Alors que des violences ont éclaté cette nuit dans certains quartiers, tout particulièrement dans les Hauts-de-Seine, j'appelle à l'apaisement. Monsieur le sénateur Pierre Laurent,

En réaction à la crise sanitaire, la France et la Suisse avaient en effet levé les restrictions fiscales et sociales qui freinaient jusqu'alors le recours au télétravail par les travailleurs concernés.

pérenne et favorable au télétravail des frontaliers. Aujourd'hui, ces derniers sont inquiets et craignent que, au-delà du 30 juin prochain, la possibilité de télétravailler soit de nouveau limitée. En décembre dernier, un accord fiscal a été conclu, leur permettant de télétravailler jusqu'à 40 % de leur temps de travail, sans modification des règles d'imposition sur le revenu. Je note cependant qu'une incertitude demeure

C'est un signal prometteur pour des milliers de frontaliers. Pour autant, la France n'a toujours pas fait part de ses intentions quant à la signature de cet accord. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les intentions de la France vis-à-vis de cet accord ?

En 2022, le groupe de travail mis en place pour rédiger un accord multilatéral avait recommandé que la période de souplesse soit prolongée jusqu'au 30 juin 2023, soit d'ici à quelques jours

et Républicain. Madame la Première ministre, hier matin, à Nanterre, Nahel, 17 ans, a été tué à bout portant par un membre des forces de l'ordre. Nous ne connaissons pas encore les circonstances exactes de ce drame, mais les images sont terribles. La lumière doit être faite, car un refus d'obtempérer ne peut pas et ne doit pas se terminer par la mort d'un jeune. Nos premiers mots vont naturellement à la famille de la victime et à sa maman. Toute mort est tragique, mais quand la victime a 17 ans et que les circonstances sont celles que l'on connaît, on peine à imaginer la souffrance des proches. Le temps du deuil doit être respecté.

Les enquêtes administratives et judiciaires doivent aboutir rapidement à la manifestation de la vérité, condition du retour au calme, mais cela ne sera pas suffisant. Dans de telles circonstances, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Je dénonce les tweets incendiaires de certains syndicats de policiers, minoritaires certes, mais néanmoins intolérables. Vous n'entendrez jamais de surenchère dans nos paroles. Madame la Première ministre, nous croyons à la police de la République, mais lorsqu'un drame comme celui d'hier se produit, c'est l'exemplarité de l'État de droit qui est remise en question et c'est aussi son autorité qui est potentiellement fragilisée. En conséquence, il faut objectivement évaluer l'application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure sur l'usage des armes et en tirer les conséquences. Il faut également reconsidérer la formation des policiers, et les moyens qui y sont alloués, tout au long de leur carrière. Face à cette tragédie, au-delà des paroles, vos réponses et vos actes doivent participer à l'apaisement que le pays attend. Madame la Première ministre, il y a urgence. La parole est à Mme la Première ministre.

Le Président de la République a dit, ce matin, la peine et l'émotion de la Nation. À mon tour, de nouveau, avec tout mon gouvernement, je veux adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Nahel et les assurer de toute ma solidarité. La justice est saisie, elle avance ; l'auteur du coup de feu est en garde à vue. Je souhaite comme chacun que la vérité puisse être faite au plus vite. Vous m'interrogez spécifiquement sur nos règles et sur la formation de nos forces de l'ordre. Vous connaissez tout comme moi, monsieur le président Kanner, leur engagement au quotidien. Policiers et gendarmes ont conscience de leur devoir d'exemplarité. Comme nous l'avons toujours dit, quand il y a une faute, les fonctionnaires ont à en répondre aussi bien dans le champ administratif que judiciaire. Des images particulièrement choquantes du contrôle de Nahel donnent à penser que le cadre d'intervention légal n'a pas été respecté. Mais seule la justice le dira et nous en tirerons, bien évidemment, toutes les conséquences. Dans l'immédiat, le ministre de l'intérieur prendra les décisions qui s'imposent à l'issue de la garde à vue. Monsieur le président Kanner, l'heure est au deuil, à l'enquête et à l'apaisement. Nous avons une exigence absolue de vérité. C'est elle qui nous permettra de surmonter les colères et de donner les réponses qu'attendent légitimement la famille de Nahel, les élus et les Français. La parole

L'inflation s'est installée durablement en France et le pouvoir d'achat des Français en subit les conséquences. Même si elle recule, le retour à un niveau de prix d'avant la guerre en Ukraine est illusoire. Nos compatriotes sont confrontés à une forte hausse des prix dans des secteurs de première nécessité. La précarité alimentaire s'installe, comme en témoignent les associations d'aide d'urgence qui ont accueilli 22 % de bénéficiaires supplémentaires depuis un an. Parallèlement, à l'heure de la réindustrialisation de la France, toutes les entreprises ont des difficultés pour recruter. Il en est de même dans le secteur public. Dans l'éducation nationale, dans la justice, dans les hôpitaux, dans l'armée, dans la police ou la gendarmerie, et dans les collectivités territoriales, les candidatures ne sont pas assez nombreuses et les postes ouverts aux concours ne sont pas pourvus. En réponse, le Gouvernement a privilégié la politique du chèque et de la prime, ou encore celle du bouclier tarifaire. Les salariés ne veulent pas de chèques distribués comme une aumône ou comme la pièce que me donnait ma grand-mère le samedi, quand j'étais enfant. Ils veulent tout simplement un salaire leur permettant de vivre correctement. La politique des primes et autres chèques pouvait se comprendre durant la crise sanitaire, mais cette réponse est désormais inadaptée. Si elle a permis de donner un coup de pouce momentané au pouvoir d'achat, elle risque, faute d'assujettissement aux cotisations sociales, de faire des travailleurs pauvres d'aujourd'hui les retraités très pauvres de demain.

pas uniquement avec des chèques, pour reprendre très précisément votre question, mais aussi avec des mesures importantes comme le bouclier tarifaire, que vous avez mentionné. En outre, depuis six mois, avec Bruno Le Maire et Roland Lescure,

Monsieur le ministre, un jeune homme de 17 ans est mort hier. Nahel a été abattu par un agent de police, à bout portant. Aujourd'hui, au nom du groupe écologiste, j'adresse pensées et condoléances à sa mère, à sa famille et à ses amis. Aujourd'hui, après une nuit de colère dans certaines villes d'Île-de-France, notre rôle doit être d'appeler au calme, au nom du respect pour le temps du recueillement à la mémoire de Nahel et au nom du respect de la justice et de la vérité. Ce matin, face aux images, le Président de la République a parlé d'un acte inexcusable et inexplicable. Inexcusable ? Sans aucun doute. Inexplicable ? Certainement pas. Oui, il y a des raisons qui ont conduit à ce drame. Nous nous rappelons les efforts que vous avez déployés, monsieur le ministre, pour combattre dans cet hémicycle toutes les propositions visant à améliorer les rapports entre la police et la population, vous montrant ainsi fidèle à votre doctrine 100 % répressive. Nous nous rappelons votre acharnement à vouloir interdire de filmer l'action de la police Et nous voyons comment, depuis des années, drame après drame, avec détermination, vous défendez la honteuse loi Cazeneuve, qui permet à la police d'ouvrir le feu sur les chauffeurs d'une voiture selon des conditions manifestement trop floues. Depuis que cette loi est en vigueur, on constate que les tirs sur des véhicules ont augmenté de 40 % par rapport aux cinq années précédentes.

Monsieur le ministre, si vous voulez que le calme revienne- ce que nous appelons de nos voeux -, il est temps de revenir sur cette loi. Combien de morts supplémentaires faudra-t-il pour que vous en preniez conscience ?

Il permet à chacune et à chacun de se réaliser par l'effort, quelles que soient son origine et sa condition sociale. J'ai toujours défendu cette valeur universaliste du sport, hier comme élu local, aujourd'hui comme sénateur. Nous sommes nombreux ici à rester fidèles à l'esprit de Pierre de Coubertin. À moins d'un an des jeux Olympiques de Paris, il me paraît essentiel de rappeler le caractère universel des valeurs du sport, car elles sont de plus en plus contestées dans notre pays. Le collectif Les Hijabeuses revendique ainsi le droit de participer à des compétitions officielles de football en portant le foulard islamique. Alors qu'en Iran des femmes risquent leur vie pour vivre sans le voile, en France, certaines se battent pour pouvoir l'imposer sur un terrain de football. Ces « hijabeuses » ont attaqué l'article 1 des statuts de la Fédération française de football, qui interdit « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. dernier, le rapporteur public du Conseil d'État a donné un avis favorable sur leurs revendications. Plutôt que de permettre une revendication religieuse sur un terrain de football, il est essentiel de préserver le sport de tout séparatisme. est le sens de la proposition de loi que j'ai déposée le 25 mai 2022. Soyons lucides : les islamistes s'engouffrent dans toutes les portes ouvertes, et le sport en est une. Madame la ministre, je ne vous demande pas de commenter une décision que la justice n'a pas encore rendue. Cependant, le Gouvernement est-il prêt à

Vous le voyez, nous sommes aux côtés des clubs, du mouvement sportif, pour faire respecter notre modèle républicain, notre modèle sportif, et pour combattre toutes celles et tous ceux qui voudraient y porter atteinte. Préserver le pacte républicain au coeur du sport : voilà notre détermination la plus absolue

Les Républicains. Madame la ministre, ce lundi, le rapporteur public du Conseil d'État s'est prononcé pour l'abrogation de l'article 1 des statuts de la Fédération française de football, qui interdit tout port de signes religieux lors de compétitions sportives, à la suite d'un recours formé par les Hijabeuses et Alliance citoyenne, collectifs qui instrumentalisent régulièrement nos institutions et nos principes républicains. Sans préjuger de la décision du Conseil d'État, nous tenons à vous faire part de notre vive inquiétude quant à cette attaque contre notre pacte républicain. Nous n'en serions pas là si votre gouvernement ne s'était pas opposé à notre proposition d'interdire le port de signes religieux lors des compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées. À plusieurs reprises, notre majorité a adopté une disposition en ce sens : en 2020,

dans le sport. Comme la Première ministre l'a rappelé hier, nous sommes et resterons intransigeants sur le respect de la neutralité du service public dans le sport jusqu'au coeur de nos équipes de France. Nous serons intransigeants sur la lutte contre toutes les formes de prosélytisme et de radicalisme. Nous serons également déterminés à garantir la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je crois que, sur tous ces points, monsieur le sénateur, nous regardons dans la même direction. La question que vous posez

madame la ministre : stop à l'hypocrisie et au manque de courage politique de ce gouvernement face à la radicalisation de certaines organisations et à la multiplication de ces dérives religieuses ! Si le Conseil d'État suit l'avis du rapporteur public, ne soyons pas naïfs, cela se traduira par une victoire pour celles qui souhaitent fragiliser, avec cette offensive religieuse, l'un des piliers de notre société et, par là même, par une défaite politique pour notre République. La réponse du Gouvernement ne peut se limiter à quelques contrôles ou à la signature de partenariats avec les fédérations. L'État doit mettre fin à cette spirale communautaire qui est à l'opposé des valeurs du sport et de la République. Madame la ministre, soutenez notre proposition de loi La parole est à Mme Christine Herzog, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, madame la Première ministre, mes chers collègues, j'associe à ma question Sylvie Vermeillet, sénatrice du Jura. En 2018, la SNCF a suspendu la liaison directe Metz-Nancy-Lyon en raison des travaux réalisés à Lyon-Part-Dieu, qui empêchaient son maintien. Ces travaux devaient durer quatre au cours duquel la patience des usagers de ce TGV a été mise à rude épreuve. À l'issue des travaux, la SNCF s'était engagée à repositionner la desserte qui, du Luxembourg à Vintimille, permettait aux usagers de gagner du temps et de réduire C'était un réel atout pour les quatre régions desservies, du Grand Est à Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), en passant par la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Or la SNCF vient de faire savoir qu'elle annulait finalement cette desserte pour la renvoyer, par tronçons, aux conseils régionaux concernés. En parallèle, elle conseille aux usagers d'utiliser la ligne TGV Metz-Strasbourg-Colmar-Dijon, celle-là même qui cible davantage la clientèle frontalière que la population française du centre des régions. Or le contribuable, qu'il soit alsacien ou lorrain, a tout autant financé la SNCF et mérite un égal accès au service public. Il est scandaleux que l'actionnaire majoritaire de la

Madame la Première ministre, comment pouvez-vous annoncer, le 24 février dernier, un grand plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour le secteur ferroviaire à l'horizon 2040 et, quatre mois plus tard, accepter la suppression de cette ligne indispensable au maillage de notre territoire ?

Le Gouvernement n'est pas resté inactif. Le ministre délégué chargé des transports a pris des engagements précis pour que cette liaison Metz-Lyon, qui passe par Nancy, puisse rouvrir. À la minute où nous parlons,

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour le groupe Les Républicains. Madame la ministre, en France, plus de la moitié des étudiants en première année de licence échouent. Dès lors, que pensez-vous de la casse organisée par Parcoursup ?

Parcoursup a renversé le bac, déjà affaibli par le contrôle continu et les notes qui varient d'un établissement à l'autre, et par l'angoisse de l'arbitraire froid de l'algorithme. On a déshumanisé cette dernière étape de la vie scolaire au nom d'un impératif technocratique. Parcoursup a également désorganisé l'année de terminale. Les élèves ont désormais cinq mois pour se préparer aux épreuves,

d'une régression pédagogique, qui aggrave les inégalités et obère les chances de réussite d'une jeunesse sacrifiée sur l'autel de Parcoursup. Madame la ministre, le 1 juin est devenu la journée nationale de l'angoisse ! Cessons cette absurdité bureaucratique pour l'accès au savoir ! Nous, sénateurs du groupe Les Républicains, demandons la création d'un véritable service public de l'orientation, dont le but n'est pas d'avoir 100 % de réussite au bac, mais d'instruire, de bien former et de mieux orienter. Cette ambition éducative est aussi humaniste.

durant de nombreuses années : l'indépendance, le pluralisme et la liberté des médias. Je veux vous dire notre inquiétude. À la faveur des concentrations économiques, qui monopolisent les médias aux mains de quelques groupes industriels et financiers, dont l'activité principale est le plus souvent étrangère à la presse, à l'information ou à la culture, se met en place devant nous un empire médiatique de propagande au service d'une idéologie qui prône la haine de l'autre. l'autre. M. Bolloré, qui étend son empire à la télévision, à la radio, à la presse écrite, au cinéma et à l'édition, qui en contrôle presque la totalité, y compris la majorité des livres scolaires,

c'est pour quand ?

l'ensemble de nos travées, à un sursaut. Dans un monde où toutes les démocraties sont menacées, où les populismes semblent triompher, l'enjeu de la liberté de la presse est vital c'est un enjeu républicain qui doit nous rassembler, un enjeu démocratique qui doit nous mobiliser. Je vous suggère de méditer cette phrase de Victor Hugo : « La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre Madame la Première ministre, Pierre Dac disait : « Il faut une infinie patience pour attendre toujours ce qui n'arrive jamais. réanimé en mars 2017 et promis par le Premier ministre Bernard Cazeneuve dans le cadre du plan de revitalisation de l'Amiénois, le barreau TGV Creil-Roissy a été formellement acté par un courrier adressé par le Président de la République à Mme le maire d'Amiens après que vous-même, madame la Première ministre, l'avez annoncé en avril 2019 lors d'une visite dans la capitale picarde. Le courrier précisait en outre le calendrier de ce chantier, en

Plus précisément, madame la Première ministre, peut-on encore avoir confiance dans la parole du Président de la République ? -Non ! Les engagements écrits des gouvernements sont-ils encore crédibles ?

les récents événements impliquant le groupe paramilitaire Wagner ne manqueront pas d'avoir des conséquences en Afrique. Le groupe est présent au Soudan, en République centrafricaine, en Libye, au Mali et au Mozambique. Wagner est devenu un outil important de la lutte d'influence russe en Afrique, en développant un panel d'activités allant de la protection des États à l'exploitation des ressources naturelles, en passant par les opérations d'information et, surtout, de désinformation anti-occidentales, essentiellement anti-françaises. Cependant, la rupture entre Wagner et le Kremlin a de fortes chances de déstabiliser les opérations de Wagner en Afrique de l'Ouest. En tant que parias soumis à la vindicte de leurs commanditaires russes, Wagner et son dirigeant Evgueni Prigojine pourraient se retrouver dans une position instable et délicate. Les activités brutales et sanglantes de Wagner sont largement financées par l'exploitation illégitime des ressources naturelles. C'est pourquoi les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions contre les activités de Wagner, qui visent à empêcher son expansion en Afrique. Dans ce contexte, il est crucial que la France agisse de manière énergique en intensifiant sa coopération avec ses partenaires africains, notamment dans le golfe de Guinée, très inquiets à la fois de la contagion terroriste et des milices incontrôlables. Monsieur le ministre, quelles conséquences vos services anticipent-ils en Afrique à la suite de la rupture de ban du groupe Wagner ? Et comment la France entend-elle réagir pour soutenir nos partenaires africains et protéger les intérêts de cette région éminemment stratégique ?

Il faut dire les choses telles qu'elles sont : Wagner n'est pas une société militaire privée ou une milice, mais un groupe criminel et mafieux, d'organisation- violence, prédation, manipulation, règlements de compte. C'est un groupe sur lequel la Russie s'appuie pour mener les actions qu'elle n'est pas capable de conduire avec son armée régulière. Wagner a établi, partout où il s'est déployé, la violation systématique des droits de l'homme comme principe cardinal de son action. Ce groupe a systématiquement renforcé la menace terroriste qu'il prétendait combattre. Que ce soit en Syrie, en Libye, au Mozambique, au Mali ou en République centrafricaine, Wagner est un véritable fléau, dont le seul objectif est de piller les richesses au détriment des États et des populations, et au prix d'exactions atroces. J'en veux pour preuve le rapport accablant des Nations unies, qui définit clairement la responsabilité du groupe Wagner dans le massacre de 500 civils à Moura, au Mali, en mars 2022. Nous ne laisserons aucun espace à cette organisation, qui n'hésite pas à recruter des criminels parmi les plus endurcis dans les prisons russes. Pour répondre concrètement à votre question, oui, nous continuerons à imposer des sanctions européennes rigoureuses

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour le groupe Les Républicains. L'année passée, l'apprentissage a atteint un niveau record, puisque plus de 800 000 contrats ont été signés. C'est une bonne nouvelle ! Toutefois, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, nombre de nos communes rurales nous alertent sur leurs difficultés à recruter. Les candidats sont nombreux, mais les financements ne suivent pas. pour l'année 2023, quelque 18 000 intentions de recrutement des collectivités ont été recensées, alors même que le budget prévu ne permet d'en financer que 10 000. En mars dernier, la circulaire relative au renforcement du recrutement d'apprentis dans la fonction publique pour les années 2023-2026

Les maires et l'ensemble des élus s'en inquiètent vivement, ainsi que les centres de formation et les maisons familiales rurales. Ce n'est pas faute d'avoir alerté le Gouvernement sur ce sujet lors des débats sur le projet de loi de finances. Pourtant, Mme la Première ministre a déclaré attendre un engagement fort des employeurs publics, espérant dépasser prochainement le million d'apprentis. Force est de constater qu'un décalage subsiste entre l'ambition affichée et les moyens alloués à terme, ainsi que la complexité du cadre juridique. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lui-même insiste régulièrement sur l'insuffisance des financements au regard des besoins. Aussi, monsieur le ministre, le Gouvernement compte-t-il revoir ses objectifs en matière d'apprentissage et réévaluer les moyens financiers à la hauteur des besoins des collectivités locales ? La parole est à M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques. Monsieur le

D'ici à quelques jours, nous signerons avec le CNFPT, que vous avez mentionné, monsieur le sénateur, une nouvelle convention pour l'exercice 2023-2025.

monsieur le sénateur- c'est le troisième élément que je voulais évoquer -, je ne veux pas m'arrêter là. Tous ensemble, nous pouvons faire de l'apprentissage une véritable voie de prérecrutement pour la fonction publique. Comment expliquer aujourd'hui que, à l'issue d'un contrat d'apprentissage d'une durée

sur les finances des collectivités locales. Voilà encore un transfert de charges qui n'est pas acceptable pour les élus locaux et qui est dommageable pour les jeunes en attente de formation ! La parole est à M. Olivier Jacquin, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

pour étudier la possibilité de raccourcir les durées des concessions autoroutières. Il écartait, de fait, les deux autres options mises sur la table par l'inspection générale des finances dans un rapport révélé par, à savoir la diminution des prix des péages et le prélèvement sur les bénéfices des sociétés concessionnaires.

Compte tenu du caractère stratégique des autoroutes, tant pour l'aménagement du territoire que pour la transition écologique des transports, et à moins de dix ans de la fin des premiers contrats, allez-vous publier la saisine et l'avis du Conseil d'État, comme vous vous y étiez engagé auprès de notre collègue députée socialiste Christine Pires Beaune, le 3 mai dernier ? Par ailleurs, quand allez-vous enfin lancer les Assises des autoroutes que vous nous promettez depuis trois mois ? La parole

pour les usagers spoliés, comme le dernier sketch des chèques-vacances l'a montré. L'État régulateur doit reprendre la main et préparer véritablement l'après-concessions ! Écrire et lancer de nouveaux contrats, c'est cinq ans de travail. Le Sénat vous le répète depuis 2020 : d'autres modèles existent. Notre groupe a proposé la création d'un établissement (Épic), Routes de France, qui gérerait l'ensemble du réseau routier national. Débattons-en enfin ! C'est dans l'intérêt des Français, des entreprises, des territoires et du climat. La parole

s'est exprimée et a annoncé sa décision de suspendre le projet FresH2 d'ici à la fin 2023, et cela pour plusieurs années, jusqu'à ce que le marché de l'hydrogène soit durablement établi. Je le rappelle, le projet FresH2 vise à développer la pile combustible à hydrogène destinée à remplacer le moteur diesel utilisé dans le transport. C'est le projet de reconversion industrielle du site Bosch d'Onet-le-Château, usine historique de fabrication des injecteurs et des bougies de moteur diesel, condamnée en 2020 par l'abandon précipité du diesel. La déclaration de l'industriel est un coup de tonnerre dans le ciel aveyronnais. Ce choix, sans explication et sans information préalables, apparaît comme une remise en cause des engagements pris auprès des syndicats, des élus locaux et de l'État. l'équipementier s'est engagé à maintenir 250 emplois reconvertis dans les technologies à hydrogène en 2028, en contrepartie de la transformation industrielle. L'annonce de Bosch est une condamnation des 250 derniers emplois. Or, monsieur le ministre, depuis cette annonce la semaine dernière, vous n'avez fait aucune déclaration Alors que la stratégie nationale hydrogène que vous défendez vise à développer les véhicules lourds propres et à construire en France une filière industrielle créatrice de 50 000 à 150 000 emplois, que fait le Gouvernement pour le développement du projet de reconversion de l'usine Bosch d'Onet-le-Château ? Que faites-vous pour les 250 emplois aveyronnais à convertir et à pérenniser ?

Vous le savez, la sortie programmée du véhicule thermique représente un vent de face extrêmement fort pour l'industrie automobile traditionnelle. Nous avons le temps, car elle est prévue d'ici à 2035, mais nous devons adapter l'appareil de production à ce nouveau défi.

J'ai échangé avec tous les élus : aujourd'hui avec vous, hier avec les députés à l'Assemblée nationale, mais aussi avec Mme la présidente de région, M. le président du département et M. le maire de Rodez. Nous sommes tous alignés nous devons nous assurer que Bosch tiendra ses engagements. Mon équipe est déjà en relation avec les organisations syndicales, mais aussi avec la direction de Bosch en France. Toutefois, vous le savez, cette décision sera prise en Allemagne. Je suis déjà entré en contact avec la direction allemande, avec laquelle j'échangerai de manière formelle dans les jours à venir.

que ce soit sur l'hydrogène ou sur autre chose. Je m'y engage devant vous. Et évidemment, j'informerai tous les élus du département et de la région de l'avancée de ces discussions. La

il dispensait un islam salafiste, notamment des prêches marqués par des propos légitimant le djihad armé, appelant à la violence, à la haine, à la discrimination et à la commission d'actes de terrorisme- excusez du peu Que cette personne en rupture avec les valeurs de la République soit retournée en Algérie, c'est tant mieux. C'est le résultat de la volonté de l'État- je salue la prise de position de ce jour, dans la presse, du préfet de région mais aussi, et surtout du courage, ainsi que de la pertinence des choix du maire d'Hautmont, Stéphane Wilmotte. Je veux saluer son courage, car il a refusé le mariage de cette personne, qui aurait sans doute empêché l'expulsion. Or, pour avoir dénoncé cette instrumentalisation du mariage par cet individu, le maire d'Hautmont s'est trouvé sous le feu de menaces, d'insultes et d'intimidations. Fallait-il, à ce propos, laisser s'organiser ce dimanche la manifestation de soutien à M. Sayah, qui n'avait pas d'autre objet que de faire psychologiquement pression sur le maire d'Hautmont ?

sont intolérables, mais les violences psychologiques le sont tout autant. Elles sont moins visibles, mais plus sournoises, plus fréquentes et tout aussi graves et insupportables. Aussi, monsieur le ministre, ma question est limpide : comment concevez-vous l'accompagnement de l'État quand les maires sont confrontés, à l'évidence, à des mariages de complaisance ou, pire, à des mariages forcés, et parfois à une forme de violence psychologique pour qu'ils les prononcent contre leur gré ? La parole

prônait un islam salafiste. Il était en lien avec une mosquée où était faite l'apologie du terrorisme. Après de nombreuses démarches administratives, comme dans d'autres affaires plus médiatiques que nous avons connues récemment, il a pu être expulsé du territoire national.

En raison de l'incohérence du recensement des logements assujettis à la taxe d'habitation, plus de 40 % des contribuables n'ont pas répondu. C'est le cas de plusieurs millions de foyers qui continuent à effectuer leur déclaration de revenus sur papier et qui n'ont même pas été informés. De ce fait, les services fiscaux viennent de leur adresser une circulaire leur demandant de se renseigner auprès d'eux ou de téléphoner à un numéro national en 08, afin de connaître la procédure à suivre. de cette circulaire sont d'une totale mauvaise foi, car des files d'attente de plusieurs heures ont été constatées pour accéder physiquement aux services fiscaux. Et même lorsqu'on le compose vingt fois de suite, le numéro national en 08 est toujours occupé. Selon les syndicats, en une seule journée, plus de 94 000 personnes ont été victimes de cette incurie. De plus, par exemple, plus de 20 000 courriers sont en attente de réponse dans les Bouches-du-Rhône et plus de 3 000 dans les Hautes-Pyrénées. Il est totalement inacceptable que, une fois de plus, les responsables du ministère des finances marginalisent ceux qui n'ont pas accès au numérique. Je vous demande donc, monsieur le ministre, pourquoi le formulaire papier prérempli n'a pas été adressé par la poste aux contribuables concernés, comme c'est le cas pour toutes les déclarations d'impôt sur le revenu lorsque les gens ne sont pas connectés à internet ?

Elle est importante pour les communes, puisque celles-ci continuent à percevoir une taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le Parlement a d'ailleurs décidé d'élargir la liste des communes qui peuvent majorer de 60 % la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Si nous voulons qu'elles reçoivent les justes recettes auxquelles elles ont droit,

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Les dépenses restantes devront donc faire l'objet d'une maîtrise encore plus stricte pour permettre le respect de la trajectoire fixée par le projet de loi de programmation des finances publiques. Or, non contents de comprimer ces dépenses,

groupe s'opposent à la création d'un tel livret. Quel

La commission a introduit un produit d'épargne réglementée destiné au financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense. C'est une bonne chose au regard du montant particulièrement élevé de l'épargne des Français. Nous sommes nombreux à avoir été alertés sur les difficultés rencontrées par notre industrie de défense, qui peine à mobiliser les financements dont elle a besoin, notamment

la décision récente de la Banque de France d'exclure l'armement des stratégies d'investissements responsables n'est pas non plus vécue comme un encouragement. Pourtant,

Si nous nous félicitons de la création, par la commission, de ce livret de souveraineté destiné au financement de l'industrie de défense, qui complète les soutiens budgétaires de l'État, tout de même y apporter quelques garde-fous. Il serait impensable que ce livret, aux objectifs louables, favorise les exportations au détriment des commandes nationales.

des députés Jacques Maire et Michèle Tabarot sur les travaux du Parlement européen en la matière. Ce dernier document fait état d'un manque de transparence inquiétant de l'État français en matière d'exportation d'armement. Le contenu du rapport annuel du Gouvernement délivré au Parlement

cet amendement suivent également les recommandations du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements adopté en 1998, qui demande aux pays membres d'accroître la responsabilité et la transparence au sujet du commerce des armes, en donnant aux parlements les moyens de contrôler la pratique des gouvernements. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de préciser davantage le contenu de ce rapport, auquel il faudrait ajouter plusieurs éléments, tels que le nombre de refus à l'exportation par pays, tout en précisant les critères de refus, les types et les quantités de matériel de guerre, ainsi que les destinataires. Quel

Un rapport est remis chaque année par le ministère des armées, mais son contenu ne permet pas aux parlementaires que nous sommes d'exercer pleinement notre mission, car nombre d'informations n'y figurent pas, ou de manière très lacunaire. Nous proposons un nouveau format de rapport, plus complet, incluant les armes légères et les petits calibres, le matériel à finalité duale et les composants d'armes. Le rapport devra aussi préciser les destinataires et les usagers finaux

M. Mickaël Vallet. L'article 27 prévoit la possibilité pour les services de l'État d'utiliser tout dispositif destiné à rendre inopérant ou à neutraliser un drone représentant une menace imminente pour l'ordre public, la défense, la sécurité nationale ou encore le service public de la justice,

afin de pouvoir y inclure les armes de lutte anti-drones les plus puissantes, telles que celles qui sont fondées sur l'utilisation de faisceaux laser à effet dirigé. C'est un objet qui nous paraît légitime, car il s'agit de matériels auxquels seules les autorités civiles et militaires compétentes doivent pouvoir recourir. J'émets donc un avis favorable.

Il s'agit de remplacer la formule « peut être interdit, limité ou encadré » par les mots « est interdit », afin de durcir

Guillaume Gontard. Cet amendement a pour objet d'encadrer les prérogatives confiées à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) en matière de cybersécurité. Selon la rédaction actuelle de l'article 32, l'Anssi peut utiliser certaines des prérogatives qui lui sont confiées, comme le blocage de noms de domaine, en cas de menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Malgré les explications des rapporteurs en commission, nous continuons à penser qu'il faut préférer à la notion de sécurité nationale, encore trop floue, celle d'intérêts fondamentaux de la Nation, comme le souligne l'éminent juriste M. Bertrand Warusfel, vice-président de l'association française de droit de la sécurité de la défense. Il n'est donc pas excessif de considérer que la protection des intérêts de la Nation constitue la traduction pénale de la mise en oeuvre de la stratégie de sécurité nationale. En effet, les principaux actes d'hostilité, de sabotage ou simplement d'espionnage intervenant dans un domaine susceptible de menacer la sécurité nationale peuvent être réprimés sur le fondement des articles 410-1 à 411-11 du code pénal. En d'autres termes, les poursuites pénales par le livre IV du code pénal sont en quelque sorte des instruments juridiques de la politique de sécurité nationale dont l'État a la charge exclusive. Sur cette base, autant préciser immédiatement dans cet article et les suivants la notion d'intérêts fondamentaux de la Nation, afin de renforcer la robustesse juridique du dispositif. Compte tenu de l'ensemble des prérogatives accordées à l'Anssi, notamment à propos de la liberté d'accéder au service de communication au public, qui est une composante de la liberté d'expression et de communication, consacrée à l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous estimons que cette sécurité juridique supplémentaire n'est pas un luxe. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement Cet amendement a été rejeté en commission, car le remplacement de la notion de sécurité nationale par celle d'atteinte pénale aux intérêts fondamentaux de la Nation n'est absolument pas adapté à la lutte contre les cybermenaces. De plus, le dispositif proposé est beaucoup plus protecteur des libertés que la notion d'intérêts fondamentaux de la Nation. J'émets

est à M. Pierre Laurent. Par cet amendement, le groupe CRCE propose de renforcer les pouvoirs de l'Anssi en matière de sanctions lorsque les éditeurs de logiciels font preuve d'une négligence intentionnelle envers leurs obligations d'informer leurs utilisateurs en cas de vulnérabilité ou d'incident affectant leurs produits. Actuellement, l'article 34 de ce projet de loi ne prévoit pas de sanctions financières spécifiques à l'encontre des éditeurs de logiciels. Nous estimons qu'il est crucial de remédier à cette lacune, afin de garantir une responsabilité adéquate des éditeurs et de prévenir les situations où des informations critiques en matière de défense et de sécurité nationale sont sciemment dissimulées à l'Anssi. Dans cette perspective, nous proposons de nous inspirer du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui établit des sanctions pécuniaires significatives en cas de violation des règles de protection des données personnelles. Nous souhaitons que des sanctions analogues à celles qui sont prévues par le RGPD puissent être imposées dans le cadre de l'article 34 du projet de loi lorsque les éditeurs de logiciels manquent délibérément à leurs obligations d'information envers l'Anssi. Nous renforcerons ainsi l'incitation des éditeurs à prendre leurs responsabilités en matière de sécurité. Cela contribuera à assurer un niveau adéquat de transparence et de coopération entre les éditeurs et les autorités compétentes. Cela jouera un rôle crucial dans la protection de nos intérêts nationaux en matière de défense et de sécurité.

faire connaître publiquement ces vulnérabilités-là. C'est une mesure qui attenterait directement à la réputation de ces éditeurs de logiciels et qui agirait donc comme une sanction très lourde, en contrepartie de la dissimulation de telles vulnérabilités.

afin d'assurer leur protection légale. Le droit en vigueur permet aux lanceurs d'alerte numérique de prévenir non pas directement l'entité concernée par une vulnérabilité quant à la sécurité de son système de traitement automatisé de données, mais seulement l'Anssi, sous peine de poursuites judiciaires. Au contraire, un hacker éthique encourt trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour avoir pénétré un système de traitement automatisé de données sans l'accord préalable de son propriétaire.

vulnérabilité affectant le produit d'un éditeur de logiciel ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité du système d'information et susceptible d'affecter significativement un desdits produits. Une telle reconnaissance du statut de hacker éthique permettrait aux personnes de bonne foi, qui découvrent une vulnérabilité,

du marqueur technique : il s'agirait ainsi des « éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique permettant de détecter une activité malveillante et d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information ». Quel est

Or les garanties prévues à ce stade ne portent pas sur le type de données traitées. S'agissant d'une question aussi sensible que la protection de la vie privée et le secret des correspondances, il n'est pas acceptable de renvoyer à un décret le soin de préciser la nature des données collectées. Il est essentiel de fixer des limites

ou fasciste au sein de nos armées. Néanmoins, chacun le sait, les militaires sont soumis à un régime disciplinaire robuste et complexe, qui est codifié dans le code de la défense.

L'intégrité, le respect, l'honneur et la loyauté à la patrie sont en effet des valeurs cardinales de notre armée. La diffusion d'idéologies antirépublicaines, racistes, voire nazies, en son sein, comme en témoigne l'enquête de, est un réel danger pour notre République. Cet amendement vise donc à interdire le recrutement dans l'armée de toute personne condamnée pour discrimination, provocation ou injure raciale, ethnique, religieuse ou sexiste, ainsi que pour le port d'emblèmes nazis ou d'autres régimes génocidaires. Nous en avons bien conscience, il s'agirait d'une exigence renforcée au regard de celle qui s'applique au reste de la fonction publique, car les militaires ne sont pas des fonctionnaires comme les autres.

Or la taxe foncière est le dernier véritable levier fiscal dont disposent les communes. Les recettes qui en découlent sont indispensables au financement des services publics locaux- entretien des infrastructures, éclairage public, voirie, collecte des déchets, équipements sportifs, etc.

en maintenant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du PIB à compter de 2025. » On ne

explication de vote. Monsieur le ministre, si vous voulez que nous poursuivions un débat de qualité, il faudrait que vous ne caricaturiez pas les positions que nous sommes amenés à prendre. Personne n'a dit ici que la fiabilité des engagements de la France et des alliances qu'elle a nouées reposait exclusivement sur l'indicateur de 2 % du PIB. Nous disons simplement qu'il en est une composante. D'ailleurs, vous n'avez pas à le nier, puisque vous reprenez vous-même cet objectif, malgré toutes les discussions méthodologiques que l'on peut avoir. Car, effectivement, il fait dépendre l'effort de défense de la conjoncture économique, récession ou croissance. Nous savons bien que ce n'est pas le seul indicateur. Comme vous le dites justement, puisque vous utilisez également cet indicateur, la seule question que nous devons nous poser est celle de la date.

insuffisant de leur redressement, l'absence d'arbitrage qui vous serait favorable de la Première ministre pour atteindre cet objectif en temps utile, à côté des objectifs physico-financiers qui sont évidemment au coeur de la loi de programmation militaire. Mais celle-ci forme un tout, et les 2 % sont aussi importants. Vous voulez les différer, nous voulons les accélérer. Le débat pour l'instant porte sur ce point.

Mais nous fixons aussi comme objectif de notre politique de défense de travailler à la relance d'initiatives de prévention des conflits et à la multiplication des accords multilatéraux et régionaux de désarmement.

en citer d'autres : « La LPM s'inscrit dans une visée stratégique plus globale, visant prioritairement la prévention des conflits, la lutte contre le surarmement et pour la multiplication d'accords multilatéraux et régionaux de désarmement. » Cette phrase n'aurait pas été inutile dans la description générale de nos objectifs. Pas de caricature ! On peut ne pas être d'accord avec l'amendement, mais il y a tout de même des idées auxquelles il faudrait peut-être prêter un peu d'attention.

l'Alliance atlantique dans le rapport annexé. Il faut d'abord rappeler ce qu'est une alliance militaire, d'une part, et ce qu'elle ne doit pas nous empêcher de faire pour défendre nos intérêts nationaux, d'autre part. Une alliance militaire défensive doit dissuader d'attaquer et nourrir l'esprit de défense collective pour rendre sa mise en oeuvre indubitable en cas d'attaque. L'allié français, dont il ne devrait même pas être besoin de préciser qu'il est loyal, sait parfaitement ce qu'implique son appartenance à l'Alliance et n'hésitera pas à en assumer les conséquences. une alliance militaire n'est pas la caporalisation des États européens par l'allié américain, encore moins en dehors du champ bien circonscrit de la solidarité défensive. Car, année après année, nous éprouvons cette difficulté à opposer nos intérêts aux États-Unis d'Amérique, qui, hors l'Otan, ne sont pas un allié au sens militaire, mais un partenaire au sens générique et, à notre grand regret, pas toujours de confiance. Écoutes téléphoniques des dirigeants français et allemands par la (NSA) sans que cela vraiment eu de suite ou fait scandale, interventionnisme agressif pour casser des fleurons industriels- je pense à Alstom et à la technique des otages économiques -, « coup de poignard »- l'expression est non pas de moi, mais de Jean-Yves Le Drian, que je cite assez rarement -dans l'affaire des sous-marins australiens qui se solde par une très malvenue visite d'État à Washington ... Ajoutons-y le choix d'un autre partenaire outre-Rhin dont nous sommes probablement le seul des deux à penser que nous formons un couple et qui se tourne pour ses importantes dépenses d'armement, comme cela a été précédemment évoqué, vers des matériels non européens. Le rapport annexé doit rappeler plus fortement que la France est une puissance pluricontinentale et l'Europe avec elle distingue la position d'alliée de celle de partenaire et doit s'autoriser avec volontarisme à coopérer plus activement au sud du tropique du cancer et le faire, comme le définissait ce grand penseur de la défense qu'est Régis Debray, « tous azimuts », et pas seulement en suivant l'aiguille indiquant le nord ou en se vivant comme allié quand il faut aussi être un partenaire offensif. La commission a donné un avis défavorable sur cet amendement, dont les auteurs semblent remettre en cause le caractère particulier des alliances de la France, tant dans le cadre de l'Union européenne que de celui de l'Otan. Bien évidemment, la France n'est en rien empêchée par son appartenance à l'Alliance de développer d'autres alliances tous azimuts. Si l'on précisait une telle chose, ce serait plutôt perçu comme une défiance à l'égard de l'Otan : cela n'est franchement pas approprié dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui remet en cause notre sécurité collective sur le sol européen. Quel est l'avis du

»- c'est factuellement vrai -« ne saurait empêcher la France, fidèle à sa tradition de Nation présente sur plusieurs continents et soucieuse de la coopération internationale entre les peuples de nourrir et développer des partenariats tous azimuts dès lors que ceux-ci servent ses intérêts

M. André Guiol. La commission des affaires étrangères a modifié l'article 7 du projet de loi de programmation militaire, notamment pour prévoir son actualisation à la fin de J'avais déposé en commission un amendement pour que l'actualisation intervienne au plus tard avant la fin du premier semestre 2027. Mes arguments n'étaient pas du tout les mêmes que ceux de la commission, qui a souhaité avancer cette actualisation en 2026 en raison d'importantes échéances électorales en 2027. Pour ma part, il s'agissait de rendre la date plus pertinente avec l'échéance mentionnée dans l'étude d'impact du projet de loi de programmation militaire, qui indique que l'actualisation « vise à proposer une réorientation de la trajectoire de ressources des effectifs pour la période 2027-2030

Elles se dérouleront dans les océans, pour plusieurs raisons. D'une part, si les frontières terrestres sont à peu près partout bien établies,

pour évaluer les menaces prévisibles à l'horizon 2035-2040 en particulier dans le domaine maritime et en lien avec notre réalité géostratégique mondiale et maritime,

L'amendement du Gouvernement vise à supprimer un alinéa issu d'un amendement du groupe CRCE qui correspondait au sentiment majoritairement exprimé au sein de la commission selon lequel le débat autour de la

Nous regrettons profondément l'absence de stratégie de relance politique en faveur d'initiatives multilatérales de désarmement, alors même que la revue nationale stratégique constate le détricotage inquiétant de tous ces accords. Au rythme actuel, la course aux armements n'est pas seulement dangereuse : elle ne sera pas supportable. Elle touche de surcroît tous les espaces communs, de l'espace aux fonds marins en passant par le numérique. Alors que l'avenir de la planète devrait commander de protéger ces espaces comme des biens communs inaliénables et démilitarisés, accepter comme une fatalité la militarisation exponentielle du monde revient à participer à la montée des insécurités mondiales. C'est pourquoi nous vous proposons de faire précéder de faire précéder notre stratégie d'anticipation des sauts technologiques dans le domaine des espaces communs de l'impérieuse nécessité d'une stratégie de désarmement, afin de montrer qu'il s'agit de notre priorité. Par ailleurs, la réponse donnée aux besoins de nos armées sera assurée par des filières industrielles duales qui devront aussi répondre aux besoins civils et de coopération. Les investissements en la matière doivent être placés sous contrôle public et appuyés par un fonds de financement stratégique de souveraineté sous contrôle démocratique. Cela permettra la mobilisation de capitaux mixtes, soumettant ainsi la stratégie industrielle aux besoins de la Nation.

C'est tout à fait le contraire, bien évidemment. De la même manière, considérer que l'export militaire reviendrait à stériliser les filières industrielles ne correspond absolument pas à la réalité de nos entreprises de la BITD, pour lesquelles les exportations sont au contraire absolument vitales. Quel est l'avis

des armes nucléaires (TNP), entré en vigueur en 1970. Il tend également à faire en sorte que la France rejoigne comme membre observateur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires Les deux questions sont liées. En effet, l'article VI du TNP engage toutes les parties « à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Le TNP est également clair au regard des obligations de la France comme des autres pays. En effet, selon l'alinéa 8 du préambule, les États parties déclarent « leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire ». Ces dispositions sont encore plus pertinentes à l'heure où les tensions internationales sont croissantes. La dégradation de la situation appelle à réévaluer notre politique de dissuasion en lien avec le respect de nos engagements internationaux, dont l'article VI du TNP, visant au désarmement nucléaire multilatéral. Adopter cet amendement serait également se mettre en cohérence avec l'engagement pris lors du dernier G7 par les États membres d'approfondir les efforts de désarmement et de non-prolifération visant à atteindre « l'objectif ultime d'un monde sans armes nucléaires En cohérence avec ces objectifs, le Tian complète utilement le régime juridique international interdisant les armes de destruction massive, ouvrant ainsi la voie à l'élimination totale de ces armes dans le monde entier. armes dans le monde entier. À l'ONU, la volonté de voir appliquer l'article VI du TNP a mené en 2016 à des discussions en vue de négocier un instrument juridiquement contraignant

Toutes les puissances nucléaires ont boycotté ce vote, mais l'ampleur de la demande internationale en la matière interdit de l'ignorer royalement comme nous le faisons pourtant depuis six ans. Pour éviter toute confusion et tout élément de langage abusif, je rappelle que les écologistes jugent impossible de procéder à un désarmement unilatéral de notre pays. C'est pourquoi nous ne demandons pas à la France de ratifier le Tian : nous lui demandons de reprendre le flambeau de la négociation internationale pour le désarmement mondial. Pour ce faire, nous voulons que notre pays rejoigne le Tian en tant que membre observateur pour pouvoir participer aux discussions des États membres qui souhaitent l'abolition des armes nucléaires. Cela nous permettrait d'obtenir des informations de première main sur les discussions et les développements relatifs à ce notamment en suivant les progrès réalisés dans l'interdiction des armes nucléaires et en étant informés des positions et des préoccupations des États parties. En tant qu'observateur, nous pourrions partager notre position tout en renforçant nos liens avec les États participants ainsi qu'avec des organisations internationales et avec des acteurs de la société civile impliqués sur ces enjeux.

beaucoup d'informations sur l'organisation de la dissuasion nucléaire dans notre pays, à tel point que j'en ai été moi-même surpris. Nous avons demandé

conventionnelle de nos forces. Ce n'est pas au moment où les discours menaçants se multiplient de la part de plusieurs puissances nucléaires, comme la Russie ou la Corée du Nord, qu'il faut se détourner de l'enjeu principal principal : la crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Je vous propose de retirer cet amendement après les informations que donnera M. le ministre.

monsieur le ministre.

Nous proposons de rappeler dans la LPM que la France, seul pays européen présent dans l'Indo-Pacifique, contribue à la défense du droit à la circulation maritime dans cette région, notamment en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, afin de préserver la paix et la stabilité de la région. La Chine entretient de nombreux conflits territoriaux avec ses voisins : Japon, Vietnam, Philippines, Malaisie et, bien sûr, Taiwan. La recrudescence des incidents observés en mer de Chine est liée à une volonté du régime de Pékin de s'approprier un espace maritime international. La situation devient très tendue, voire angoissante pour les pêcheurs vietnamiens, régulièrement menacés par les garde-côtes chinois. Les sénateurs philippins nous ont expliqué au Sénat que le petit récif philippin baptisé « Julian Felipe » est devenu un bouillon de tensions, depuis que Pékin le revendique comme son bastion et y a construit des des bases militaires sur des îlots artificiels. Les incursions chinoises en mer des Philippines sont désormais quotidiennes et font la une des journaux locaux. Les revendications chinoises sous les formules d'« eaux chinoises historiques », de « zones de souveraineté incontestable » et de « zones de pêche chinoise traditionnelles » ont été invalidées en juillet 2016 par des décisions du tribunal arbitral international constitué sur l'initiative des Philippines. Pékin juge la sentence « nulle et non avenue ». Non content de ne pas respecter le droit international quand il n'est pas conforme à ses objectifs, Pékin menace directement la libre circulation du commerce international, en affirmant que les eaux du détroit de Taïwan sont sous souveraineté chinoise. Cette approche prédatrice de la Chine, associée à une marine de guerre qui progresse en nombre, crée l'escalade. Elle est même susceptible de déclencher un conflit international si Pékin rompt le en tentant d'envahir Taiwan, à l'image de ce que nous observons en Ukraine avec la Russie. Voilà pourquoi il est important que la France défende le droit à la circulation maritime.

les conclusions du rapport d'information adoptées à l'unanimité par notre commission s'appuient sur un travail de fond qui ne peut pas être modifié ici sans une discussion approfondie avec les rapporteurs.

Or nos rapporteurs ont entendu sur place les autorités se plaindre, lors de leur audition, de ne pas avoir été informées, par exemple, du passage d'un Rafale en Nouvelle-Calédonie. L'évolution récente de la situation de la Polynésie française souligne, si besoin était, que la méthode appliquée jusqu'ici ne renforce peut-être pas suffisamment le lien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. La rédaction issue du rapport d'information sur la place de la France dans l'Indo-Pacifique, qui a été adopté- je le rappelle -à l'unanimité, tente de remédier à cette situation. Elle s'appuie sur un travail de fond, et nous ne pouvons pas la modifier comme cela en séance.

» Ayant été ministre des outre-mer, je ne peux pas être suspecté de débarquer complètement dans cette affaire. Je vais d'où cela provient ! Les familles politiques indépendantistes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie demandent cette cogestion. Je l'ai refusée à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de cogestion en matière régalienne dans notre Constitution entre une collectivité territoriale à droit spécifique et le coeur même de notre souveraineté qu'est le modèle d'armée

Nous proposons donc la suppression du passage qui y fait référence. Nous souhaitons également que, outre les réservistes, les élèves des établissements scolaires occupent une place importante dans les cérémonies commémoratives.

remet au Parlement un rapport au 1 octobre 2023 faisant état d'un bilan du SNU préalablement à toute évolution du dispositif.

Nous vivons aujourd'hui une crise de recrutement des enseignants, qui sont d'ailleurs particulièrement opposés à ces missions. Je ne crois donc pas que nous pourrons compter sur eux. Enfin, la jeunesse s'engage ; nous en avons la démonstration tous les jours. Appuyez-vous davantage sur les collectivités locales, pour voir comment on peut associer